La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 28 mai 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure, présentée par MM. Jean-François Husson, Vincent Segouin, Mme Catherine Dumas et plusieurs de leurs collègues

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans cette France du 2 juin 2020 qui retrouve le goût et le plaisir de la liberté, j'ai l'honneur de présenter cet après-midi à notre Haute Assemblée un texte attendu et espéré : une forme de réponse à tous les chefs d'entreprise, qui, dans l'ensemble des territoires de notre République, ont appelé les pouvoirs publics La crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore a été d'une violence inouïe, sans précédent, par l'ampleur des victimes humaines qu'elle a causées et par le choc économique qu'elle provoque. Face à la vague épidémique, les mesures prises par les pouvoirs publics ont été inédites. Jamais dans notre histoire récente nous n'avions vu un pays si brutalement mis à l'arrêt- d'ailleurs, près de la moitié de la planète -, et l'ensemble des établissements, à l'exception de quelques-uns nécessaires à la vie quotidienne, fermés sur décision administrative. Cet arrêt brutal de l'économie a fort logiquement entraîné des pertes importantes, voire colossales pour les entreprises, subitement privées de demande alors que l'appareil productif se redressait depuis quelques années. Nos entreprises ont fait face à un effondrement de leurs marges et à une baisse de chiffre d'affaires sans précédent, quand elles n'étaient pas tout privées de chiffre d'affaires, tout en devant honorer leurs charges. Des emplois sont aujourd'hui menacés et la hausse du chômage, rendue publique la semaine passée, est un sujet de préoccupation majeure. Face à cette situation économique, la réaction logique des entreprises a été de se tourner vers leurs assureurs, pour pouvoir, à côté des mesures de soutien de l'État, bénéficier de leurs garanties.

Il n'aurait pas été anormal d'avoir une réactivité plus forte, plus rapide, plus puissante, en allant- c'est ce qui s'est passé plus tard

je ne partage pas cette vision défaitiste de l'action publique. Comme nous avons souhaité le rappeler dans l'exposé des motifs de notre proposition de loi, des « obligations morales » s'imposent aux compagnies d'assurance, pour intervenir et soutenir les entreprises face à des événements exceptionnels, auxquels nous n'avions jamais été confrontés. Il y avait donc urgence à sortir de l'impasse en se hissant à la hauteur des enjeux : c'était une question de survie économique. Cette crise a d'ailleurs permis de souligner le rôle et l'importance du politique et de la puissance publique. Nous aurions en effet manqué à nos responsabilités et, d'une certaine manière, à la confiance des Français si nous n'avions pas proposé rapidement de nouvelles solutions. Une première réponse de court terme a été apportée par l'État, avec l'indemnisation du chômage partiel, extrêmement généreuse, et les reports de charges, bientôt transformés en annulations. Les nombreux chefs d'entreprise que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon département m'ont témoigné de l'importance de ces mesures pour la survie de leur activité. Mais, nous le savons- le débat a eu lieu telles mesures ont un coût particulièrement important pour nos finances publiques et il n'est pas « philosophiquement » souhaitable que la totalité des dispositifs de soutien revienne à l'État. Avec mes collègues parlementaires Catherine Dumas et Vincent Segouin, et soutenus par plus de 150 des nôtres, nous avons jugé nécessaire de faire des propositions rapidement, au plus fort de la crise, pour brosser le contour de solutions nouvelles. Nous l'avons bien senti, le modèle sur lequel la relation entre les compagnies d'assurance et les entreprises est construite ne pouvait pas fonctionner dans le cadre d'une crise d'une telle ampleur. Nous avons donc pensé qu'il fallait innover, en partant des besoins des entreprises et en instaurant un dialogue nourri avec les assureurs. La proposition de loi que nous vous présentons a trois objectifs : tirer les leçons du passé en instaurant un nouveau dispositif garantissant un niveau de protection équivalent pour toutes les entreprises entreprises ; définir les responsabilités respectives des assurances, de l'État et des assurés pour éviter que ne se reproduisent les querelles actuelles ; présenter un partenariat nouveau et original associant l'État et les assureurs pour assurer conjointement et solidairement dans les faits la protection de nos entreprises contre les événements sanitaires exceptionnels. En quelque sorte, nous avons cherché à créer un « paratonnerre économique » reposant sur la responsabilité partagée entre l'État et les assureurs. Quatre principes fondent ce nouveau dispositif. Premièrement, les assurances couvriront obligatoirement toutes les entreprises contre les événements sanitaires exceptionnels

Sans dimension obligatoire, il y a le risque d'une insuffisance de l'assiette des cotisants. Celles qui pourraient se permettre de s'en passer ne seraient plus dans la communauté d'intérêts des acteurs économiques. Deuxièmement, le financement du risque est assuré par une cotisation additionnelle au contrat, qui permettrait de constituer des provisions pour les assurances. Elle viendrait abonder un fonds d'État, d'État, instaurant une forme de solidarité entre les assurances pour l'indemnisation des entreprises touchées. Notre proposition de loi prévoit pour ce fonds un abondement annuel minimal de 500 millions d'euros. Troisièmement, l'indemnisation des entreprises est possible dès lors que les mesures prises pour lutter contre une crise sanitaire entraînent des pertes de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. 50 %. Quatrièmement, pour indemniser les entreprises victimes de la crise, les assurances seraient aidées par le fonds d'État au des indemnités à verser.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme vous le savez, la présente proposition de loi est au coeur d'une actualité brûlante qui fait la une de nos journaux depuis le début de la crise sanitaire. Dès les premières mesures de confinement et de fermeture des lieux publics, la question de la mobilisation des assureurs pour soutenir nos entreprises a déchaîné les passions. En dépit des engagements pris par le secteur assurantiel, le constat réalisé au début de la crise a été sans appel : les assureurs ne sont pas au rendez-vous. cette absence s'explique par le caractère difficilement prévisible et « systémique » de l'épidémie, qui en fait un risque inassurable. Néanmoins, par le passé, le législateur est déjà intervenu pour remédier aux lacunes des garanties offertes par les assurances. Ainsi, en 1982, après les terribles inondations de 1981, la loi a défini un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. C'est pourquoi il nous revient aujourd'hui d'être force de proposition pour répondre aux attentes de nos entreprises, qui se tournent vers l'État mais aussi vers les assureurs, afin de traverser ces moments difficiles. Aujourd'hui, alors que la crise sanitaire laisse la place à une crise économique profonde et durable, l'examen de cette proposition de loi nous permet de poser les jalons d'une future couverture assurantielle. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a instauré un groupe de travail associant l'État, la Fédération française de l'assurance (FFA), les entreprises, des parlementaires, dont notre collègue Jean-François Husson, pour mener une réflexion sur le sujet. Avant d'aborder le contenu de la proposition de loi, je tiens tout d'abord à saluer le travail effectué par Jean-François Husson et les coauteurs, qui, en quelques semaines seulement, sont parvenus à élaborer un dispositif complet, nous permettant d'avoir un débat riche aujourd'hui. La tâche était particulièrement ardue ; les auditions que j'ai menées ont souligné à quel point la conciliation des intérêts de chacun constituait un véritable « château de cartes Pour les entreprises, l'enjeu est évidemment de garantir une couverture juste, tout en contenant le montant de la prime. Pour les assureurs, il s'agit de délimiter le dispositif, afin de pouvoir absorber le montant des indemnisations à verser. Pour l'État, l'objectif est de protéger le tissu économique, de préserver la stabilité du secteur assurantiel et de limiter le coût pour les finances publiques. Pour parvenir à une solution équilibrée, les paramètres à définir sont très nombreux le fait déclencheur, le champ de l'indemnisation, le périmètre des entreprises bénéficiaires, le montant des primes, le mode de déclaration et de versement de l'indemnisation, la présence d'une franchise, les conditions de mobilisation du fonds et son abondement, ainsi que les conditions de réassurance publique. Chacun de ces facteurs modifie l'équilibre financier du dispositif. Ce n'est pas très simple ... L'appréciation budgétaire de ce mécanisme, en particulier de son coût pour les entreprises, est d'autant plus difficile que le groupe de travail constitué par le ministère commencerait tout juste à réaliser de premières projections financières. Cette absence de recul nous encourage aujourd'hui à une certaine prudence dans la construction de notre jugement. En tant que rapporteur, j'ai souhaité examiner ces dispositions avec un triple objectif : préparer l'avenir pour éviter les divergences auxquelles nous avons pu assister entre les assureurs les assureurs ; sécuriser nos entreprises en leur permettant de passer un cap de trésorerie difficile ; garantir un partage équilibré des responsabilités et des coûts entre les assurés, les assureurs et la solidarité nationale. J'en viens désormais à l'examen des cinq articles de la proposition de loi. Le premier article prévoyait initialement l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à l'application de mesures administratives en cas de crise sanitaire. Cette assurance prend la forme d'une garantie obligatoire des contrats d'assurance contre les dommages d'incendie souscrits par les entreprises, ce qui permet une large couverture des assurés et une simplification. Cette garantie est couverte par une cotisation additionnelle. Le Le dispositif proposé est très protecteur, à double titre. D'une part, l'ensemble des entreprises sont concernées, sans distinction de statut juridique, de taille ou de chiffres d'affaires. D'autre part, les entreprises bénéficiaires sont à la fois celles dont les pertes d'exploitation résultent directement des mesures administratives en vigueur, comme les restaurants, avec la fermeture des lieux de confinement, et celles dont les pertes sont indirectes.

La principale porte sur la notion même de pertes d'exploitation. En effet, il m'a semblé que la philosophie du dispositif était davantage de sauvegarder temporairement une entreprise pour lui permettre de passer ce cap difficile, en la soulageant de ses charges fixes,

L'indemnisation des pertes d'exploitation serait colossale en cas de crise systémique comme celle de la Covid-19, ce qui serait de nature à renchérir le coût de la prime pour les entreprises. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement visant à indemniser les charges fixes de l'entreprise, plutôt que ses pertes d'exploitation, dès lors qu'elle subit une baisse de chiffre d'affaires, ou

La commission a également adopté deux autres amendements visant à rendre le dispositif efficace pour les entreprises, en permettant un versement rapide à l'entreprise et en encadrant par voie réglementaire le montant de la prime. Elle a aussi précisé le champ des mesures administratives permettant de déclencher cette garantie. garantie. L'article 2 crée un fonds alimenté par un prélèvement obligatoire acquitté par les assureurs et assis sur les primes des contrats d'assurance de biens professionnels. Ce fonds contribue à l'indemnisation des charges fixes. La commission a adopté un amendement tendant à préciser la vocation de ce fonds. Ainsi, ses ressources ne sont décaissées que dans le cas de crise sanitaire grave. Pour les menaces ou risques sanitaires d'une ampleur contenue, il peut être considéré que les assureurs mutualisent les primes reçues et indemnisent les entreprises sans faire appel au fonds. En d'autres termes, ils font leur métier. Il s'agit de poser une double exigence envers les assureurs, en leur demandant d'assurer un risque financé par des cotisations additionnelles et, en plus, de participer à un fonds servant de « réserve de précaution » pour les crises sanitaires majeures. Cette configuration présente un double intérêt. D'une part, elle permet de pérenniser les ressources du fonds, car, s'il avait été sollicité pour l'indemnisation du moindre sinistre, ses ressources disponibles n'auraient pas permis de faire face à une crise d'ampleur nationale, en particulier si son financement ne repose que sur les assureurs. D'autre part, ce schéma permet de garantir une forme de « ticket assureurs », c'est-à-dire qu'il leur revient d'assumer une part du risque. En effet, si les assureurs avaient seulement perçu des primes pour les verser au fonds, leur rôle aurait été réduit à celui d'un « collecteur Ce dispositif à plusieurs vitesses est renforcé par le mécanisme de réassurance publique prévu à l'article 3. Si les assureurs ne peuvent faire face au montant des indemnisations à verser, la Caisse centrale de réassurance peut jouer son rôle de réassureur. Elle bénéficie de la garantie de l'État, permettant à ce dernier d'intervenir en tout dernier ressort si besoin. Mes chers collègues, comme je l'ai indiqué lors de l'examen en commission, je ne puis que souscrire aux objectifs de cette proposition de loi ; je l'avais d'ailleurs Elle nous donne aujourd'hui l'occasion de nous prononcer en faveur d'une première « architecture assurantielle » et de déterminer les responsabilités de chacun dans la mise en oeuvre de ce « paratonnerre économique », pour reprendre la formule des auteurs du texte. Nous avons souhaité jeter les bases d'un schéma de partage des risques entre les entreprises, l'État et le secteur assurantiel. Nous devons néanmoins garder à l'esprit que le mécanisme a vocation à évoluer au cours de la navette. Il devrait également pouvoir être enrichi à mesure que les services de l'État mais aussi les entreprises du secteur assurantiel parviennent à modéliser plusieurs scénarios et à évaluer le coût de cette nouvelle garantie pour les entreprises. La parole

l'épidémie que nous traversons est un événement qui n'a pas d'exemple dans notre histoire récente. Ses conséquences économiques sont encore difficiles à chiffrer précisément, mais nous sommes certains d'une chose : elles sont massives.

le 13 avril dernier. Parce que de telles crises pourront se reproduire à l'avenir, il est nécessaire de créer un régime de type assurantiel destiné à intervenir en cas de future catastrophe sanitaire majeure.

toutes les parties prenantes, afin de rendre concrète l'idée d'un régime assurantiel spécifique. Je tiens d'ailleurs à remercier les élus, dont les sénateurs Jean-François Husson et Michel Raison, qui participent activement à ce groupe de travail sur l'assurance des risques exceptionnels. Les échanges sont riches en contenu, constructifs dans l'esprit et transparents dans la forme. Déjà quatre séances ont eu lieu ; elles ont permis de s'interroger sur les principaux paramètres d'un futur dispositif de couverture des risques exceptionnels destiné aux entreprises : la typologie de dispositif et de contrat, le champ des périls à couvrir, la délimitation des événements déclencheurs, les modalités d'indemnisation, les schémas de partage des risques. Plusieurs options sont à l'étude sur chacun de ces thèmes, et le travail se poursuit. Un thème fait néanmoins l'unanimité. Les enjeux financiers associés aux risques à couvrir sont colossaux et nécessiteront de trouver des solutions de remplacement à une solution assurantielle habituelle, à moins d'imposer à nos entreprises une charge qui serait démesurée. En effet, selon des estimations préliminaires, la Fédération française de l'assurance évalue à 120 milliards d'euros le coût théorique des pertes d'exploitation pour une durée de confinement de deux mois, ou environ 50 milliards d'euros hors salaires et bénéfices. Cette somme est à rapporter aux primes annuelles d'assurance dommages aux biens professionnels collectées, qui s'élèvent à environ 4,5 milliards d'euros. Je crois que la différence parle d'elle-même. Or ce sont ces primes qui permettent de provisionner un risque futur. De plus, un dispositif associé à une surprime de 12 %, à l'image du régime des catastrophes naturelles, permettrait de récolter annuellement environ 540 millions d'euros de surprimes annuelles, ce qui correspond à peu près au montant de toutes les primes des contrats pertes d'exploitation en France, de l'ordre de 600 millions d'euros aujourd'hui.

poursuivre les travaux et trouver ce mécanisme supplémentaire au mécanisme assurantiel classique. Nous avançons vite : sur la base des discussions qui seront finalisées dans les prochains jours, le groupe de travail rendra ses conclusions à la mi-juin. Il proposera un nombre réduit de scénarios, qui feront ensuite l'objet de plus larges consultations avec toutes les parties prenantes durant l'été. Cela permettra d'aboutir d'ici à la rentrée à un dispositif opérationnel pouvant répondre aux attentes de nos concitoyens. Je remercie le sénateur Jean-François Husson de cette proposition de loi. C'est une manière de prendre date. Cela pourra constituer la première pierre d'un édifice qui devra être consolidé dans les prochaines semaines. Je souhaite en effet que nous trouvions une traduction législative définitive dans le courant de cette année pour ce mécanisme assurantiel de protection des entreprises face à des crises majeures. il nous reste à finaliser les consultations techniques auprès de toutes les parties prenantes sur la base des scénarios dessinés par le groupe de travail avant que la représentation nationale ne poursuive ses travaux. Si la présente proposition de loi met en avant des principes auxquels nous souscrivons et qui répondent aux attentes des élus, comme la simplicité, l'accessibilité et l'indemnisation rapide, je n'aurai pas la présomption de dire que nous disposons aujourd'hui tous les éléments pour cristalliser les contours exacts et précis du dispositif. Je suis certaine que le groupe de travail saura proposer une ou plusieurs solutions d'assurance offrant une indemnisation satisfaisante aux entreprises pour un coût acceptable tant pour les entreprises assurées que pour l'État. Le dialogue et le travail vont donc se poursuivre. Notre débat aujourd'hui en est une étape importante. Je sais que nous pouvons compter sur l'entière coopération des élus durant cette période, afin de trouver ensemble un dispositif pertinent, utile et durable. Il y va de la résilience à venir de nos entreprises et de notre capacité à résister collectivement aux chocs futurs. La parole

ont participé, d'abord un tout petit peu, puis, sous la pression, de plus en plus. Nous nous réjouissons donc de voir examiner par la Haute Assemblée une proposition de loi de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure. Le texte qui

à hauteur de la totalité des sommes économisées du fait de la diminution importante des sinistres, nous nous sommes dit qu'un texte plus global, incluant cette ambition contributive,

leurs capacités financières et des dividendes qu'ils partagent régulièrement. Depuis le début de la crise, la question de l'engagement des assureurs s'est posée

ne plus attendre la pression des opinions publiques et les demandes des élus. Il faut faire en sorte que les contributions des assureurs soient immédiates et organisées. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il est pour nous extrêmement important

La crise sanitaire du Covid-19 a révélé les carences de la couverture assurantielle des entreprises pour les pertes d'exploitation ne résultant pas d'un dommage. En effet, comme l'ont avancé les assureurs, le risque de pertes d'exploitation n'est pas couvert par la plupart des contrats d'assurance souscrits par les entreprises, du fait de son caractère facultatif, mais aussi parce qu'il doit être rattaché à un dommage matériel comme un incendie ou un bris de machines. Dans la crise actuelle, il est cependant naturel que Dans la crise actuelle, il est cependant naturel que les assureurs participent à l'effort de solidarité nationale. C'est en tout cas un avis largement partagé par le Président de la République, le Gouvernement, de nombreux parlementaires de toutes sensibilités et les entreprises, petites ou grandes. Cette participation est moralement d'autant plus justifiée que, du fait de la crise sanitaire et des mesures administratives de confinement prises par le Gouvernement, le niveau de sinistralité des compagnies d'assurance a fortement chuté pendant plus de deux mois pour les principaux risques de dommages. La Fédération française de l'assurance chiffre cette économie à environ 300 millions d'euros par mois, ce qui représenterait aujourd'hui un total de l'ordre de 750 millions d'euros.

Ces économies, dont le fait générateur est une décision administrative, me semblent très largement sous-estimées par les compagnies d'assurance. L'on sait que le total annuel des indemnisations au titre des dommages s'établit à environ 40 milliards d'euros, soit 3,3 milliards

Compte tenu de ces éléments, l'économie réelle est certainement de trois à cinq fois le montant annoncé par la Fédération française de l'assurance. Sous la pression, le secteur s'est engagé à verser 200 millions d'euros au Fonds national de solidarité en faveur des petites entreprises et des indépendants, mise qui a été doublée quelques semaines plus tard pour tenter de répondre aux critiques du Gouvernement et du Parlement, en particulier du Sénat. Je voudrais rappeler que, fin avril, lors du PLFR 2,

Ce feuilleton, qui ne me semble pas encore définitivement clos, me laisse perplexe, surtout lorsqu'une grande organisation professionnelle revendique un effort de 3,2 milliards d'euros,

Cette situation, que l'on peut déplorer, a été un élément de motivation important pour l'émergence de cette proposition de loi, tout comme elle explique les délais dans lesquels nous sommes amenés à l'examiner.

face à une crise sanitaire d'envergure et de proposer des solutions relativement simples, comme son caractère obligatoire et son rattachement à la couverture du risque incendie. Je pense que nous pouvons encore améliorer ce texte en prenant en compte certains amendements.

Rapprocher ce dispositif du critère d'éligibilité au Fonds de solidarité ne me paraît pas justifié, car, dans ce dernier cas, il s'agissait d'une subvention d'un montant forfaitaire limitée, plutôt destinée à faire passer un cap difficile aux petites entreprises en termes de trésorerie.

aurait par ailleurs le mérite d'être plus conforme aux approches habituelles des compagnies d'assurance en termes de couverture des pertes d'exploitation. Examinant ce texte dans une certaine urgence, nous n'avons pas, à mon sens, suffisamment de recul sur la crise économique qui s'annonce, notamment son impact sur les pertes d'exploitation effectives des entreprises. Sur le principe, nous approuverons toutefois cette proposition de loi, en remerciant ses auteurs de leur initiative et en espérant que la navette parlementaire et la poursuite du dialogue avec les différentes parties prenantes permettront de la compléter et de l'améliorer.

paye la même prime que lui. Comment intégrer les efforts pour faire face à l'urgence écologique dans le calcul des assurances ? Alors que les assurances reposent sur un risque quantifiable, donc assurable et mutualisable, comment modéliser les pandémies,

nous examinons cet après-midi la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure. majeure. Le texte qui nous est proposé n'est pas sans rappeler les termes de la demande formulée par le directeur général d'Axa il y a quelques semaines dans la presse, visant à créer après la crise du coronavirus un régime d'assurance pandémie. En effet, dans son interview du dimanche 5 avril dernier, général d'Axa, M. Thomas Buberl, avait annoncé sa volonté de « créer après la crise du coronavirus un régime d'assurance pandémie inspiré de celui qui existe déjà pour les catastrophes naturelles et qui pourrait appartenir à 50 % à l'État et à 50 % à un pool d'assureurs privés ». Or, il se trouve que la proposition de nos collègues ambitionne, selon l'exposé des motifs, d'« instaurer une couverture obligatoire des entreprises par les assurances pour les pertes générées par une menace ou une crise sanitaire grave », mais aussi « de permettre le financement de cette couverture obligatoire par un fonds L'analogie entre les propos du directeur général d'Axa et l'exposé des motifs est assez frappante. Nos collègues sont suffisamment rigoureux pour connaître les besoins des entreprises, qui subissent les conséquences des fermetures et des baisses d'activité. Je rappellerai ici les propos de la présidente de la Fédération française de l'assurance, qui, le 13 avril dernier, déclarait au : « En France, les pertes d'exploitation liées à la pandémie se chiffrent à près de 60 milliards d'euros. Si nous devions indemniser l'intégralité des pertes d'exploitation, cela reviendrait à mettre le secteur de l'assurance à terre. » Pourtant, ces dernières années, le chiffre d'affaires du secteur de l'assurance a progressé en France, au point de placer l'Hexagone en tête du marché européen, avec 2 609 milliards d'euros de cotisations. Sans doute sera-t-il nécessaire, à un moment, d'établir un bilan exhaustif et sincère de l'intervention des assurances auprès des entreprises dans cette crise. Ainsi, l'assureur français numéro 1 a enregistré un bond de 80 % de son bénéfice net, à 3,86 milliards d'euros en 2019, étant versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Et on demande en même temps aux salariés de prendre entre 5 et 10 jours de congés payés au mois d'avril ... Alors, quand on parle de mettre en place un « paratonnerre économique qui protégerait les entreprises des pertes d'exploitation consécutives à une menace, il semblerait que la couverture proposée ne soit pas tout à fait intégrale. En réalité, les petites entreprises ne paieront pas forcément la surtaxe demandée sur leurs contrats pour les protéger contre les pertes d'exploitation générées par les mesures prises dans le cadre d'une menace ou d'une crise sanitaire grave. À l'inverse, il est prévu que l'État prenne en charge les salaires avec le chômage partiel, les impôts et les taxes. 13 avril dernier, le Président de la République déclarait, dans son allocution télévisée : « Les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. pour que les compagnies d'assurance s'engagent à verser dans un premier temps 400 millions d'euros pour l'hôtellerie-restauration dans le plan Tourisme, alors même que, sur la période, la diminution mécanique du nombre d'accidents a permis aux assureurs d'économiser plus de 2 milliards d'euros d'indemnisations. C'est d'ailleurs toute la subtilité de cette proposition de loi, qui semble critiquer l'absence « morale » des assureurs, mais qui fait financer la garantie uniquement par les entreprises et l'État. Puisque la proposition de loi appelle les compagnies d'assurance à la générosité, sous la forme d'une contribution au Fonds d'indemnisation des très petites entreprises, je rappelle que les 400 millions d'euros initiaux versés par les assurances pour aider l'hôtellerie-restauration représentent moins de 1 % du total des réserves des assurances, qui se sont élevées en 2019 à 54 milliards d'euros. Ces résultats vont probablement augmenter en 2020, puisque, selon l'UFC-Que Choisir, le confinement a entraîné une chute de 91 % des accidents corporels, et par conséquent diminué les indemnisations des compagnies d'assurance pour un montant compris entre 1,4 milliard d'euros et 2,3 milliards

travaillé. Le risque existe, avec ce modèle, que seules les grandes entreprises aient les reins financiers assez solides pour prendre cette garantie. En cas de nouvelle crise sanitaire, elles seront indemnisées par leur assurance.

Cette proposition risque donc d'être d'une efficacité assez limitée, les petites entreprises étant aussi celles qui sont le plus fortement soumises aux divers aléas. Si elles ne peuvent obtenir une indemnisation de la part de leur assurance, elles seront comme aujourd'hui contraintes de demander l'aide de l'État ou éventuellement de cesser complètement leur activité. Enfin, cette proposition est, selon nous, encore trop déséquilibrée, puisqu'elle exige des pouvoirs publics de prendre en charge les dépenses de personnel, les impôts et les taxes tout en laissant les grandes entreprises bénéficier des aides de leurs assurances et maintenir le cas échéant le versement des dividendes aux actionnaires. Compte tenu

la théorie des hasards consiste à réduire tous les événements du même genre à un certain nombre de cas également possibles et à déterminer le nombre de cas favorables à l'événement dont on cherche la probabilité Ainsi le mathématicien Laplace définissait-il, voilà près de deux siècles, la discipline alors novatrice du calcul des probabilités. Le langage est clair, net, précis. Clair, net et précis, au point de laisser croire que l'esprit humain serait capable de réduire le hasard à des nombres, capable d'identifier tous les possibles de ce monde, capable, enfin, d'épuiser l'imprévu par le seul usage de la raison. Or l'imprévu a la fâcheuse habitude de ne jamais se présenter tel qu'on l'attendait. Il se réinvente sans cesse. Il excède toujours le cadre que nous croyions avoir taillé à sa mesure. Tel a été le cas avec la crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement. Elle nous oblige à considérer un risque nouveau, celui d'une épidémie généralisée, qui bloque d'un coup le pays tout entier. Mais il faut distinguer les facteurs qui ont provoqué la crise sanitaire de ceux qui ont provoqué la crise économique. La crise sanitaire tient à la propagation fulgurante d'un nouveau virus particulièrement dangereux. La crise économique tient au choix politique que nous avons fait pour y répondre. Nous avons choisi de privilégier la santé à l'économie. Si le Gouvernement n'a pas hésité à faire ce choix, le Parlement n'a pas non plus hésité à le soutenir dans ce choix. Je le dis, car d'autres pays, confrontés à une situation similaire, ont fait des choix opposés. L'avenir dira si la crise économique se révèle pour eux moins sévère. Le présent atteste déjà que la crise sanitaire les frappe plus durement. Le choix que nous avons fait est probablement le bon. Nous ne devons pas en douter, mais nous devons l'assumer, avec ses conséquences. Les dommages subis par nos entreprises dans cette crise s'avèrent d'ores et déjà colossaux. Mais ces dommages, parce qu'ils relèvent justement de ces décisions inédites que nous avons prises, n'entrent pas dans les cases actuellement prévues par notre droit. Comme nombre d'entre vous, mes chers collègues, j'ai été interpellé par des acteurs du territoire et des professionnels de l'assurance, dès le début du confinement. Ils ont vite pris conscience du choc économique qui les attendait. Nombre d'entre eux étaient au désespoir- je pèse mes mots -, car ils refusaient de choisir entre le sens patriotique, qui leur commandait de participer aux efforts du pays contre le virus, et leur conscience professionnelle, qui les enjoignait de ne pas manquer à leur poste malgré les risques sanitaires. Au reste, ils croyaient déjà avoir la solution à ce dilemme. Cette solution, c'est la police d'assurance, qui permet précisément la couverture contre un risque. Charge à l'assureur, ensuite, d'affronter l'imprévu s'il se présente. D'où l'incompréhension des Français au début de la crise : comment se peut-il que les assureurs, dont le métier consiste justement à anticiper les risques et accompagner les particuliers face aux imprévus, n'aient pas couvert les pertes d'exploitation subies par nos entreprises ? Comment se peut-il qu'ils n'y aient pas été tenus par des obligations contractuelles ? C'est là le signe que le cadre assurantiel n'est pas adapté et que l'état d'urgence sanitaire doit encore être amélioré pour bien lutter contre une pandémie. C'est là le signe, pour le législateur, qu'il faut agir et changer la loi. Je me réjouis donc que le Sénat se soit rapidement emparé de ce sujet. Plusieurs propositions ont été mises sur la table, et nous discuterons ensemble des différentes options. Avec mes collègues du groupe Les Indépendants, j'ai déposé le 8 avril une proposition de loi visant à créer un mécanisme d'assurance des pertes d'exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves. Je l'ai dit, il s'agit d'articuler deux logiques : d'une part, la santé, qui impose la solidarité nationale ; d'autre part, l'économie, qui impose la responsabilité individuelle. Le mécanisme que nous devrons choisir aujourd'hui devra trouver un point d'équilibre entre ces deux logiques. La solution que j'avais proposée consistait ainsi en un mécanisme d'assurance contre les pertes de recettes ouvrant droit à un crédit d'impôt. Il revêtait à mes yeux deux avantages : le premier, c'est qu'en restant à l'initiative des entreprises il mettait les acteurs privés en situation de responsabilité le second, c'est que, par l'incitation, il faisait participer la solidarité nationale à cette responsabilité individuelle. Je parle déjà au passé, car je crois que nous devons agir vite. Je sais le travail sérieux qu'a fait la commission des finances, sous la houlette du rapporteur et de l'auteur de la proposition de loi, que je tiens à le saluer. Leur proposition a déjà recueilli de nombreux soutiens. je ne crois pas utile, à ce stade des discussions, de remettre en question le principe même du dispositif. Cependant, je suis convaincu que nous pouvons encore l'améliorer lors de nos échanges. Je vous soumettrai plusieurs amendements en ce sens, qui visent notamment à préciser les modalités de calcul de la baisse d'activité dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et à faciliter la reprise d'activité pour les entreprises assurées. Mes chers collègues, alors que les Français vivent à plein le déconfinement, on pourrait facilement dire que nous nous y prenons un peu tard. Je crois pour ma part qu'au contraire nous nous y prenons très tôt : l'objectif qui nous rassemble est non pas de faire une loi de circonstances pour la crise actuelle, mais bien de poser un cadre pour pouvoir à l'avenir agir efficacement, si d'aventure nous étions amenés à décider d'un nouvel état d'urgence sanitaire. la Barca disait que « le pire n'est pas toujours certain ». Mais c'est parce que le pire n'est pas toujours certain que nous devons sans cesse renouveler nos efforts pour l'éviter. Notre responsabilité consiste aujourd'hui à élaborer le meilleur dispositif, en espérant

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les débats que nous avons eus à l'occasion de l'examen du deuxième projet de loi de finances rectificative ont bien montré toute l'étendue des interrogations que suscite, en cas de crise sanitaire grave, la question de la contribution des assurances à l'effort de maintien du tissu économique et de redressement du pays. Ces débats nous ont également montré les insuffisances et les lacunes du droit existant en la matière. C'est dire si le sujet que nous traitons aujourd'hui est capital, alors que la pandémie que nous traversons est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue notre pays depuis la grippe espagnole il y a un siècle. Nous tenons donc à saluer l'initiative prise par Jean-François Husson et ses collègues de présenter cette proposition de loi : elle vise à définir en pareille circonstance les rôles respectifs du secteur des assurances, d'une part, et de la solidarité nationale, d'autre part, dans le soutien aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, bref au tissu économique et social dans tous les territoires de France. Nous savons bien que les compagnies d'assurance enregistrent, malgré elles, des résultats exceptionnels sur la couverture des dommages. Il aura pourtant fallu qu'elles soient sous le feu des critiques de leurs assurés et sous la pression du Gouvernement et du Parlement

l'une visait à relever la taxe sur les excédents des provisions des sociétés d'assurance ; l'autre, adoptée sur l'initiative du groupe Union Centriste, proposait d'appliquer une taxe exceptionnelle de 10 % sur la réserve de capitalisation des assureurs. Mais le Gouvernement ayant indiqué conduire des négociations avec le secteur des assurances, nous avons bien voulu renoncer à ces mesures par la voix de notre rapporteur général en commission mixte paritaire. Madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous indiquer où en sont vos pourparlers sont vos pourparlers et où en est le plan d'investissement d'un milliard d'euros annoncé en concertation avec la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner les entreprises dans un plan de relance et sur le long terme ? ? La perspective, déjà proche, d'un troisième collectif budgétaire pourra-t-elle aboutir à une solution satisfaisante pour tous ? J'en viens maintenant au coeur de la proposition de loi qui n'a évidemment pas vocation à s'appliquer de manière rétroactive. Au contraire, l'assurance relative aux crises sanitaires que propose ce texte ne vaudrait que pour l'avenir, dans l'hypothèse où surviendrait une nouvelle crise d'ampleur. loi a donc pour objectif de bâtir un cadre pérenne, sans qu'il soit nécessaire de colmater les brèches dans l'urgence par voie d'amendements au gré des budgets rectificatifs. C'est donc un texte d'importance qui a vocation à dépasser les seules circonstances immédiates pour s'inscrire dans le temps long avec, en toile de fond, la préservation en cas de grave crise sanitaire du tissu entrepreneurial et productif français. Le texte contient deux volets qui nous semblent opportuns et complémentaires : créer une couverture obligatoire des entreprises par les assurances pour les pertes générées par une menace ou une crise sanitaire grave ; corrélativement- c'est important -, permettre le financement de cette couverture obligatoire par un fonds, mutualisé entre les assureurs et abondé par l'État. L'examen du texte en commission des finances a permis de l'enrichir substantiellement et je tiens ici à saluer le travail de notre rapporteur, Claude Nougein. Premièrement, plutôt que de calculer l'indemnisation sur les pertes d'exploitation, comme le prévoyait la mouture initiale du texte, la commission propose de la fonder sur les charges fixes de l'entreprise. Cela permettrait à la fois d'approcher ses coûts fixes et de ne pas renchérir inconsidérément le coût de la prime pour les entreprises. Deuxièmement, le calibrage du dispositif nous semble lui aussi parfaitement cohérent, en ce qu'il réserve l'octroi de la garantie aux seules entreprises les plus en difficulté et selon des critères d'éligibilité comparables à ceux de l'actuel fonds de solidarité. notre commission a apporté des modifications au texte en ce qui concerne le montant des primes payées par les entreprises. Elles devront faire l'objet d'un encadrement par voie réglementaire de façon à prémunir les entreprises contre toute dérive dans la fixation des tarifs. toujours dans une même logique d'efficience, la commission des finances a souhaité préciser les délais de versement des indemnisations aux assurés. Le texte initial de la proposition de loi comportait quelques écueils que le travail du rapporteur a permis de gommer afin que les entreprises soient très rapidement indemnisées, ce qui est évidemment essentiel en pareille circonstance. Concernant la création du fonds de soutien de l'État proposé à l'article 2, la mutualisation entre les assureurs des ressources destinées à l'indemnisation, d'une part, et la contribution de l'État à ce fonds, d'autre part, constituent deux points forts qui me paraissent importants. Par sa composition et sa structure, ce fonds d'indemnisation permettra opportunément de limiter le montant de la prime versée par les entreprises. Enfin, la clarification apportée par la commission concernant le rôle dévolu à ce fonds, recentré sur les crises de grande ampleur, à l'image de celle que nous connaissons, nous apparaît là encore totalement justifiée. En conclusion, c'est sans la moindre réserve

pour m'étonner du passage très éphémère dans notre hémicycle de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, qui nous a quittés au bout de trente minutes. J'avais cru comprendre que le ministre auquel elle est rattachée attache beaucoup d'importance au sujet que nous traitons aujourd'hui et je pense que les professionnels qui nous écoutent pourraient être surpris de cette attitude. mes chers collègues, nous vivons une période inédite de l'histoire de notre démocratie. Jamais un gouvernement n'avait décidé de stopper son économie et contraint sa population à se confiner et à renoncer à sa liberté de circulation. Face au risque pandémique, la France a fait le choix de la quarantaine. Ce choix, inédit, d'un confinement général et non ciblé a imposé à un nombre considérable d'entreprises et de commerçants de fermer, les privant pendant deux mois de toute ressource financière. Cette situation revêt un caractère encore plus prégnant à Paris, une des premières destinations touristiques mondiales où se concentre un grand nombre de commerces- je pense notamment aux restaurants. Cet épisode catastrophique pour le secteur touristique parisien et français en général vient s'ajouter à une succession dramatique, depuis plusieurs années, d'événements inédits dans leur ampleur et leur enchaînement et qui n'ont eu de cesse de malmener les restaurateurs, les hôteliers, les entreprises touristiques- je pense bien sûr aux

Les professionnels se sont naturellement tournés vers leurs assurances pour que leurs pertes d'exploitation soient prises en charge. Leurs demandes ont souvent été refusées par les assureurs au motif que les pandémies n'étaient pas couvertes par les contrats d'assurance, y compris par les contrats multirisques. Cette réaction des sociétés d'assurance a provoqué, outre la colère des assurés, outre la colère des assurés, une interrogation légitime dans notre pays : à quoi servent les assurances si elles ne sont pas au rendez-vous quand une entreprise voit son activité compromise en raison d'un événement, dont elle n'est évidemment pas responsable ? L'étonnement des acteurs concernés était d'autant plus grand que les pertes d'exploitation liées à une catastrophe naturelle sont couvertes. Il existe des assurances santé ou décès, des assurances pour couvrir un événement reporté ou annulé, des assurances facultatives contre le risque de pertes d'exploitation liées à une épidémie-

Il existe en réalité une différence importante entre une catastrophe sanitaire et une catastrophe naturelle. Cette dernière est directement responsable des dommages causés par un événement naturel imprévisible. Dans le cas d'une catastrophe sanitaire, ce n'est pas celle-ci qui entraîne directement des dommages, en l'espèce les pertes d'exploitation,

une clause particulière qui prévoyait une indemnisation du préjudice constitué par les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative. Au même titre que la clause « meurtres ou suicides dans l'établissement », le tribunal a décidé que cette clause particulière s'appliquait dans le cas d'une fermeture administrative consécutive à un risque sanitaire. Par ailleurs, sous la pression médiatique, plusieurs sociétés d'assurance ont accepté de prendre en charge une partie des pertes d'exploitation, sans que le contrat les y engage, dans une démarche extracontractuelle solidaire. Nous nous en félicitons. Cependant, pour la plupart des entreprises, la couverture n'existe pas. La clause d'Axa concerne seulement 10 % des restaurateurs assurés. Il convient donc de créer un nouveau dispositif assurantiel. La présente proposition de loi vise à préparer l'avenir et ne peut répondre directement à la situation actuelle de manière rétroactive. Néanmoins, ses auteurs, Jean-François Husson, Vincent Segouin et moi-même, estimons- nous l'avons précisé dans l'exposé des motifs -qu'il incombe au secteur des assurances un devoir moral d'intervention et de soutien pour compenser, autant que possible, les pertes financières des entreprises assurées. Le dispositif que nous proposons consiste à créer une cotisation additionnelle des entreprises à leur contrat obligatoire de protection de leurs biens contre l'incendie afin de financer le risque de pertes d'exploitation en cas de menace ou de crise sanitaire grave. Cette nouvelle garantie assurantielle protégera l'ensemble des entreprises, y compris celles qui subissent des pertes financières indirectes, comme les hôtels qui n'ont pas été contraints de fermer par les autorités,

d'un minimum de 500 millions d'euros par an alimenté par un prélèvement obligatoire acquitté par les assureurs, dont le taux sera fixé chaque année par voie réglementaire et assis sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance des biens professionnels. Les pertes d'exploitation seront donc prises en charge financièrement à la fois par les entreprises à travers les primes qu'elles acquitteront et par les assureurs eux-mêmes à travers un prélèvement. Enfin, nous avons prévu que la Caisse centrale de réassurance puisse pratiquer des opérations de réassurance des pertes d'exploitation consécutives consécutives aux mesures prises en cas de menace ou de crise sanitaire grave avec la garantie de l'État, si jamais les assurances ne peuvent pas faire face financièrement. Sous l'impulsion de son rapporteur, notre collègue Claude Nougein, dont je tiens à saluer la qualité d'écoute la commission des finances a modifié plusieurs points du texte initial. Nous agréons ces modifications, qui visent avant tout à limiter le coût assurantiel pour les entreprises. il a été décidé de supprimer la notion de pertes d'exploitation pour la remplacer par celle de charges fixes. En effet, la proposition de loi a pour objet non de sauvegarder les bénéfices, mais de sauver l'entreprise- cela a été dit plusieurs fois, mais je crois que c'est le message le plus important. le personnel, les assurances n'ont pas besoin de couvrir quelque chose qui est déjà pris en compte par le dispositif de chômage partiel. Réduire le champ de la couverture permettra de limiter le montant de la cotisation additionnelle pour les entreprises. Cela permet également de supprimer la franchise pour les entreprises, puisque l'indemnisation sera calculée en fonction des coûts fixes. Toujours dans l'objectif de limiter le coût de la prime pour les entreprises, la garantie ne s'appliquera

Par ailleurs, la commission a prévu quatre niveaux d'intervention en fonction de la gravité de la situation : en premier, l'assureur ; en deuxième, le réassureur ; en troisième, le fonds d'indemnisation créé par la présente proposition de loi ; en quatrième, l'État.

et, s'agissant du secteur de la restauration, de leur permettre de continuer d'incarner l'art de vivre à la française, tellement apprécié dans le monde entier..

souscrits par les entreprises et examiner la présence de clauses prévoyant l'indemnisation de pertes d'exploitation dans les circonstances de la crise du Covid-19.

que la prise en compte de la perte de chiffre d'affaires est évaluée sur la période de crise sanitaire, ce qui constitue un lien de concomitance, non de causalité.

mesures. Quel est l'avis de la commission ? en effet, l'alinéa 4 de l'article 1 précise déjà que la baisse de l'activité économique doit être consécutive à l'application des mesures administratives en question. Par ailleurs, l'amendement pourrait être plus restrictif pour les entreprises que le texte de la commission et avoir des conséquences non voulues par leurs qu'il pourrait être interprété comme limitant le bénéfice de l'assurance aux entreprises, dont l'activité est expressément visée par ces décisions administratives. Or nous avons souhaité une rédaction qui englobe à la fois les entreprises qui subissent des pertes directement liées aux décisions administratives et celles qui ont des pertes indirectes. Par exemple,

Il convient de prolonger cette période d'une période « post-crise », durant laquelle l'activité des entreprises assurées peut poursuivre sa tendance largement au-dessous du chiffre d'affaires habituel ou reprendre en forte augmentation. le présent amendement vient au soutien des assurés ; dans le second, il modère l'aide aux entreprises au bénéfice des assureurs. ? L'objet de cet amendement s'éloigne de la logique assurantielle et traite plus largement de la question du soutien à la reprise de l'activité des entreprises. La philosophie du dispositif assurantiel que nous proposons est de permettre de sauvegarder temporairement les capacités productives de l'entreprise qui ne peut fonctionner normalement. Au-delà de la période d'application des mesures extraordinaires, si la reprise n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas à l'assureur de l'assumer.

Par ailleurs, tout accroissement du de l'indemnisation renchérira également le coût du régime et le montant des primes qu'il conviendra de collecter pour en assurer l'équilibre financier. Nous demandons le retrait de cet amendement. Monsieur Decool,

Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à exclure du bénéfice de l'indemnisation les charges variables d'exploitation, qui peuvent être ajustées au sein de l'entreprise, pour ne conserver que les charges fixes. Cela semble plus équitable, de nombreux éléments pouvant entrer dans le calcul des charges variables. Quel est l'avis de la commission ?

du compte de résultat. Par ailleurs, il tend à supprimer une précision inutile afin de permettre, en cas de changement de mode de financement, de ne pas avoir à modifier l'article L. 125-8 du code des assurances.

ou une cotisation additionnelle calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté. Cet amendement a pour objet de préciser que l'assiette du taux est assise sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent et, pour les nouvelles entreprises, sur un montant forfaitaire de chiffre d'affaires fixé par arrêté.

la cotisation ne peut pas être assise sur le chiffre d'affaires, parce que cela est très variable selon le type d'entreprise. Ensuite, c'est un remboursement de charges fixes et non pas de chiffre d'affaires. Il s'agit du taux de la prime et pas du taux d'indemnisation. Retrait ou, défaut, avis défavorable.

Je partage pleinement l'objectif de cet amendement, sans aucun doute. Ce point avait d'ailleurs été soulevé lors des auditions que j'ai menées. Nous avons tous en tête la crise sanitaire actuelle, qui s'étale sur plusieurs mois, et c'est sûrement la raison pour laquelle vous avez souhaité que plusieurs versements puissent être effectués à l'entreprise. à l'entreprise. Toutefois, nous ne pouvons préjuger l'ampleur des crises sanitaires futures et des besoins des entreprises. Nous pourrions tout autant avoir une crise encore plus grave,

par l'Unédic dans le cadre du chômage partiel. Je pense que c'est un excellent rythme, et c'est peut-être plus sécurisant pour les entreprises.

doit intervenir dans un délai de trente jours après la date de fin d'application des mesures prises en cas de menace ou de crise sanitaire. À défaut, l'indemnisation sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Le porter à 8,15 % me semble exagéré et pourrait nuire à la solvabilité des assureurs. Il faut tenir compte des montants colossaux des indemnisations à verser aux entreprises.

permettant la répartition des ressources du fonds est pris après avis d'une commission interministérielle, qui est chargée de se prononcer sur l'ampleur des indemnisations dues aux assurés. Je souhaite que cet avis soit pris auprès des acteurs du fonds,

Ensuite, l'arrêté n'a pas besoin d'un avis conforme d'une autorité, étant donné que les critères de mobilisation du fonds sont objectifs et prévus par l'article. Nous avons décidé de créer une commission interministérielle, qui est consultée au moment du décaissement des ressources du fonds et qui a pour vocation d'organiser une discussion entre les acteurs du secteur assurantiel pour faire le point en cas de crise sanitaire grave.

du Gouvernement ? Les modalités de fonctionnement et de financement du fonds d'indemnisation créé à l'article 2 de cette proposition de loi soulèvent un certain nombre de questions, notamment sur le niveau de sa dotation financière, qui doit être suffisant pour assurer la prise en charge des sinistres mentionnés à l'article 1. Toutefois, sans préjudice de notre analyse globale sur ce dispositif, l'intervention d'une commission interministérielle pour le seul besoin de mobiliser les ressources d'un fonds d'indemnisation semble injustifiée. L'amendement permettant d'alléger la procédure envisagée, nous y sommes favorables.

ce qui entraînerait une charge de trésorerie importante pour les assurances. De plus, l'amendement vise une date mentionnée à l'article L. 125-11 du code des assurances : il s'agit de la date de réception par l'assureur de la déclaration de sinistre. On ne comprend pas comment une date propre à chaque indemnisation peut être commune à tous les assureurs. L'idée est plutôt que l'assureur fasse une déclaration unique auprès du fonds pour l'ensemble des sinistres dont il a la charge, plutôt qu'une déclaration par sinistre. Retrait

pour communiquer à la Caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu'ils sont amenés à verser. Ce délai me semblant assez court, je souhaiterais le porter à soixante jours.

La prescription biennale concerne les actions qui portent sur la validité, la nullité ou l'exécution du contrat. Ce sont, par exemple, les actions en responsabilité engagées contre l'assureur. Heureusement, d'ailleurs, que les assurés ne disposent pas d'un délai de deux ans pour déclarer un sinistre.

aboutirons-nous à un dispositif proche dans sa conception, c'est-à-dire avec un fonds, une prime, le rôle de l'État précisé. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Cependant, faute de temps, faute de temps, nous n'avons fait aucune audition. C'est quand même rare de déposer et de voter un texte sans aucune audition. Je rappelle que, lorsque le Sénat avait travaillé, notamment, sur les catastrophes naturelles ou sur d'autres textes, il y avait eu une mission d'information, puis une proposition de loi et un travail d'un an.

n'y a pas d'urgence. D'ailleurs, c'est bien parce qu'à un moment donné il y a eu des embouteillages, si je puis dire, aux urgences, avec un certain nombre de personnes qui ont fini par y laisser leur vie, que la panique s'est emparée

voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure. Mes chers

Il ne vous aura pas échappé que la portée de la présente proposition de loi a grandement évolué par rapport à son objectif initial, tel qu'il était exprimé dans la première version de ce texte, que j'avais déposé en mars 2017. Cet objectif n'était ni plus ni moins que de faciliter et de sécuriser le recours aux procurations électorales. La procuration, si elle déroge effectivement au principe constitutionnel du secret du vote, n'en demeure pas moins, lorsqu'elle est correctement employée, un outil indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie moderne. N'oublions pas que, déjà dans l'Athènes de Périclès, tous les citoyens ne pouvaient en pratique se rendre quotidiennement sur la Pnyx pour voter ; la démocratie en souffrait. À présent, dans une époque où notre société devient toujours plus complexe, et alors qu'elle est confrontée à une crise sanitaire inédite, l'usage de la procuration prend tout son sens. Il doit donc être rendu aussi effectif que possible. Faciliter l'acte de vote est un impératif démocratique ; c'est notre rôle, en tant que parlementaires, que d'en faciliter l'établissement. Certains obstacles s'opposent pourtant actuellement à cet exercice effectif.

cette solution intuitive, elle avait probablement aussi l'immense qualité de faciliter la vie de l'administration en évitant l'envoi d'un courrier recommandé au mandataire. Malheureusement, cela revient surtout à laisser nombre d'électeurs dans le flou. Il arrive ainsi régulièrement que le mandant oublie de notifier le mandataire de l'établissement de la procuration. Dans cette situation, bien que le mandant ait établi la procuration dans les règles, il perd son vote. encore, dans l'éventualité où plusieurs personnes établiraient des procurations au bénéfice d'un seul mandataire sans que ce dernier soit informé de l'ensemble de celles-ci, ce qui est également chose courante, seule la première demeurera valable. Dans ce scénario, il serait possible que le mandataire ignore l'existence de l'unique procuration qui soit effectivement valable. Le choix de renoncer à l'information automatique du mandataire a donc créé un angle mort administratif aussi superflu qu'ennuyeux. Y remédier était à l'origine l'objet principal de ma proposition de loi. Je l'avais déposée à nouveau en octobre dernier. À cette époque, le Covid-19 n'avait pas encore fait son apparition à Wuhan. Depuis, les événements que nous connaissons tristement bien se sont produits. Le déroulement des élections municipales de mars 2020 a été grandement perturbé ; leur second tour a été reporté à la fin du mois de juin.

C'est dans le cadre de ces travaux que les présidents Bas, Retailleau et Marseille ont déposé, le 22 mai dernier, une proposition de loi visant à mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020. L'objectif de ce texte était de contribuer à parvenir à un équilibre entre, d'une part, l'impératif de protection de la santé de nos concitoyens, et, d'autre part, la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des institutions démocratiques municipales. repousser les élections n'est pas une décision à prendre à la légère. Du point de vue des principes, cela serait relativiser la fixité et la périodicité des mandats. Du point de vue pratique, cela contribuerait à ralentir l'investissement public local, au moment même où l'économie est en grande souffrance.

voulaient faire en sorte que les pouvoirs publics soient informés de la situation sanitaire par le conseil scientifique suffisamment en amont pour que, le cas échéant, un report en bon ordre du scrutin demeure possible.

Toutefois, un tel texte n'aurait pas pu être inscrit à l'ordre du jour à temps pour les élections. Dès lors, la commission des lois a choisi d'employer ma proposition de loi comme véhicule législatif de ces mesures. J'approuve pleinement la direction qu'a prise la commission dans son travail, sous la houlette de son rapporteur, François-Noël Buffet, dont je salue l'excellent travail. Je défendrai tout à l'heure plusieurs amendements visant à préciser certaines dispositions du texte dans l'esprit qui avait été celui de mon projet initial. L'un d'entre eux a pour objet d'inscrire de manière pérenne dans le droit l'article 1 tel qu'il sera éventuellement amendé par mes propositions.

Je propose également que les autorités compétentes informent systématiquement de la procuration, par voie électronique, la préfecture de département du mandataire. Celle-ci en informerait à son tour, également par voie électronique, la commune du mandataire.

Cette disposition permettrait également à un mandant de donner procuration jusqu'au jour du scrutin en cas d'empêchement soudain. Dans les faits, cette faculté était souvent inopérante du fait du délai d'acheminement.

L'autorité administrative qui se déplace est parfaitement capable de juger de la volonté du mandant et de sa capacité à donner mandat à un tiers. J'en veux pour preuve le fait que, lorsque l'autorité considère le mandant inapte, elle n'établit pas la procuration.

Là encore, l'autorité compétente est parfaitement en mesure de constater qu'une personne ne peut pas se déplacer. En conclusion, j'espère qu'en adoptant cette proposition de loi le Sénat enverra un signal aux

m'adresser ici au Gouvernement : au cours des derniers mois, il nous a démontré sa capacité à faire preuve d'une grande célérité pour l'adoption de ses projets de loi, pourtant bien plus longs et complexes que cette modeste proposition de loi. Espérons que cet activisme ne se limite pas aux seuls textes omnibus portant habilitations Jadis, Jacques Coeur avait adopté pour devise : « À coeur vaillant, rien d'impossible ! » Je ne peux donc que vous inciter, monsieur le secrétaire d'État, à faire preuve de vaillance sur ce texte sénatorial, dont l'adoption finale n'a rien d'impossible ! La parole

pour désigner les conseils municipaux de 4 857 communes de toutes dimensions, dont certaines des plus grandes de France. Ce scrutin a fait l'objet de beaucoup d'incertitudes ; il y a quelques semaines encore, nous étions en plein confinement et personne n'imaginait qu'on pourrait le tenir. Le Gouvernement a finalement décidé de convoquer les électeurs, par un décret pris mercredi dernier ; nous sommes maintenant sur la voie de l'élection. Il n'empêche que beaucoup de nos concitoyens sont anxieux à l'idée de s'exposer à la promiscuité dans les bureaux de vote, malgré toutes les mesures d'organisation qui pourront être prises ; d'autres, sont particulièrement vulnérables, ont été malades, ou sont encore affaiblis par la maladie, hésitent à se rendre aux urnes. Nous souhaitons qu'ils aillent mieux d'ici au 28 juin, mais il nous paraît tout à fait essentiel que des mesures soient prises pour les rassurer. Nous comptions le faire en parfaite harmonie avec le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, car cela répond, de notre point de vue, qui est un point de vue républicain,

beaucoup de réactions positives, y compris dans les rangs de la majorité de l'Assemblée nationale, pourrait aboutir en temps utile. Pour cela, encore eût-il fallu que le Gouvernement déclenchât la procédure accélérée,

Mais le Gouvernement, alors même qu'il ne s'est pas opposé aux dispositions que nous proposions, n'a pas mobilisé cet instrument constitutionnel.

-la certitude que cette volonté de bien faire fonctionner la démocratie au cours du scrutin du 28 juin n'est pas partagée par le Gouvernement, puisqu'il n'a pas mobilisé les moyens nécessaires pour que le régime des procurations soit assoupli Monsieur le secrétaire d'État, vous allez vous en expliquer. Peut-être trouverez-vous que mon propos est excessif ; si tel est bien le cas, je le retirerai, bien sûr ! Peut-être avez-vous songé à d'autres instruments que la procédure accélérée qui nous permettraient tout

ne pourra pas être adopté dans un délai qui permettrait d'organiser l'assouplissement du régime des procurations. C'est donc un mauvais cheval qu'enfourche ce cavalier ; le seul bon cheval, c'est le nôtre

des élections municipales de 2020, personne n'a jamais mis en cause la légitimité de la majorité parlementaire. Eh bien, on ne doit pas non plus mettre en cause la légitimité des maires lorsqu'ils sont élus avec un faible taux de participation ! Pour autant, je crois qu'on doit à la République et à la démocratie de faire en sorte que les électeurs puissent largement se mobiliser pour exprimer un choix. on l'a bien vu pendant cette crise, où les communes ont été extrêmement réactives, tout comme les départements et les régions, le rôle des communes aura été extrêmement important tant pour gérer l'épidémie que pour en sortir et permettre la reprise

et que l'organisation des bureaux de vote présente toutes les garanties nécessaires pour prévenir les risques de contamination ; enfin, nous voulons nous assurer que le dépouillement se déroulera dans des conditions qui garantissent la sécurité sanitaire de ses opérations.

-, mais simplement pour défendre la libre expression du suffrage universel en donnant à nos compatriotes les moyens de voter, même lorsqu'ils ont peur de sortir de chez eux.

Gestes barrières » et « distanciation physique » : autant d'expressions que nous ne connaissions pas, ou à peine, il y a six mois et qui font aujourd'hui partie prenante de notre quotidien. Vous le savez, en annonçant, le 22 mai dernier, la décision d'organiser le second tour des élections municipales dans les presque 5 000 communes où le premier tour n'avait pas été conclusif, le Premier ministre a agi en conscience et en responsabilité. En conscience, parce que cette décision a été prise sur le fondement de l'avis du conseil scientifique et après avoir consulté élus et formations politiques. En responsabilité, parce qu'elle est assortie d'un certain nombre d'obligations, tant pour la campagne que pour à assurer le respect des gestes barrières, mais aussi parce que cette décision est réversible au cas où la situation sanitaire l'exigerait. En ce moment même, d'ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale examine un projet de loi qui doit nous préparer à cette éventualité. dit, dans ce contexte et comme nous y a invités le rapport du comité scientifique du 18 mai dernier, nous devons garder à l'esprit plusieurs éléments.

ensuite, nous devons faire tout notre possible pour favoriser la mobilisation des électeurs, diminuer l'abstention et nous assurer que tous ceux qui le souhaitent puissent voter.

S'agissant de l'élection à proprement parler, nous interviendrons bien, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, pour assouplir le régime des procurations, pour élargir les cas où un délégué peut se déplacer, supprimer la nécessité d'un motif pour établir une procuration et permettre à ces délégués de recueillir des procurations dans des lieux ouverts au public.

Qu'il s'agisse des mesures portant sur les procurations ou de celles qui concernent l'organisation des opérations de vote, nous avions réussi à les mettre en place dans des délais restreints avant le premier tour. Nous avons aujourd'hui un mois devant nous pour nous préparer au mieux, de manière conjointe entre État et communes, comme nous l'avons toujours fait.

pas. Il n'est d'ailleurs pas défavorable à la mesure centrale de ce texte, consistant à porter à deux le nombre de procurations qu'un même mandataire peut détenir. Si le Parlement souhaite procéder à cette évolution pour le second tour des élections municipales du 28 juin prochain, en raison de l'état d'urgence sanitaire et du contexte épidémique que nous continuons de connaître, le Gouvernement soutiendra évidemment ces initiatives.

Au demeurant, la présente proposition de loi, dont le Gouvernement partage l'ambition- faciliter l'exercice du vote -, pose certaines difficultés qu'il faut savoir souligner. devoir informer le mandataire qu'une procuration a été établie à son nom ferait porter une charge lourde et importante sur les fonctionnaires de police et les maires. Cela reviendrait sur l'avancée qu'a permise un décret de février 2004- 2004- Nicolas Sarkozy était alors ministre de l'intérieur -, qui prévoyait la fin de l'obligation d'information du mandataire. Son objet était d'affirmer qu'il revenait à la personne qui établissait une procuration d'en avertir son mandataire, et non aux pouvoirs publics. Cette position du ministre de l'intérieur de 2004 nous paraît toujours pertinente. Elle traduit, surtout, le fait que cette règle ne relève pas du niveau législatif, puisqu'il avait alors été procédé par décret.

les maires qui vérifient qu'un mandataire n'est pas porteur de plus d'une procuration. Or qu'en est-il ? L'Insee n'est techniquement pas en mesure de permettre cette vérification, qui vise à limiter le fait qu'une même personne détienne des procurations

mais aussi de la suppression du motif justifiant le recours à la procuration. C'est également le cas des dispositions relatives au matériel mis à la disposition des électeurs pour assurer leur protection lors du vote. Le ministre de l'intérieur s'y est déjà engagé : non seulement nous retiendrons toutes les préconisations du conseil scientifique, mais encore l'État prendra à sa charge l'équipement des bureaux de vote dans les communes, partout où cela sera nécessaire.

notamment après l'annonce de la fermeture des écoles, des collèges, des lycées et des universités, puis des bars et des restaurants, et à l'instauration de mesures de confinement. Il faut dire que

tour. Pour les conseils municipaux qui n'ont pas été élus ou qui ne l'ont pas été au complet en mars, lesquels représentent une minorité de communes, mais une large majorité des électeurs inscrits, le scrutin a été fixé au 28 juin.

de faciliter, voire de promouvoir les procurations, car cela permettra de gagner quelques points de participation et de satisfaire un nombre non négligeable d'électeurs, notamment de personnes âgées.

organiser les élections municipales rapidement, dans de bonnes conditions, et installer les exécutifs locaux. Tout cela relève d'un impératif moral, politique, cela a été dit, mais aussi démocratique, économique et social.

27 mai. J'ai l'habitude d'être aimable, particulièrement avec mes collègues, mais aussi honnête intellectuellement. Que dire donc de l'article 2 , qui prévoit la mise à disposition des équipements de protection nécessaires à la sécurité sanitaire ?

le maintien du premier tour des élections municipales quarante-huit heures, je le rappelle, avant l'annonce du confinement total du pays. L'exécutif a décidé de maintenir le premier tour en sachant pertinemment que le second ne pourrait avoir lieu comme prévu.

Les personnes âgées et les parents de jeunes enfants ont été les premiers abstentionnistes « contraints » du premier tour. Le second tour s'annonce tout aussi sombre. La vague de chômage- le nombre de chômeurs a augmenté de 843 000 en avril -est significative de la détresse dans laquelle vont se retrouver un grand nombre de Françaises et de Français.

régime démocratique est malade, mes chers collègues, et ce depuis longtemps. Nos institutions sont minées par le présidentialisme et le néolibéralisme.

aujourd'hui que par son impuissance. Elle favorise le développement d'un régime autoritaire d'exception, alors qu'elle pourrait accoucher d'une République des communs, plus juste, plus égalitaire, plus participative. La campagne électorale pour le second tour ne pourra pas se dérouler dans les conditions habituelles garantissant une proximité avec les électrices et les électeurs. Le manque de lisibilité de l'organisation du scrutin du 28 juin et l'impératif de sécurité des opérations électorales font douter de la portée réelle des propositions dont nous débattons aujourd'hui. Les enjeux vont bien au-delà des seules questions techniques.

les procurations électorales, introduites en 1946, ont longtemps été réservées à certains électeurs. Leur périmètre s'est peu à peu élargi, notamment après la suppression du vote par correspondance en 1975. Aujourd'hui, elles servent à remédier à l'absence temporaire d'un électeur, pour des raisons tant personnelles que professionnelles. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi vise à améliorer l'information du mandataire, en précisant qu'il est informé de la demande d'établissement de la procuration et des conditions d'organisation du vote.

À cet égard, je regrette la suppression du volet « mandataire » du formulaire de procuration depuis 2006. Plus largement, la proposition de loi vise à sécuriser les opérations de vote. Le jour du scrutin, et jusqu'à la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote et les représentants des candidats seraient chargés de contrôler la régularité des procurations. Je me félicite de ce que ce dispositif n'ait pas été conservé par la commission, de la régularité des procurations établies relevant du maire, sous le contrôle du juge de l'élection. Il n'appartient pas au bureau de vote de refuser d'enregistrer le vote d'un mandataire et de contrôler la compétence territoriale de l'autorité devant laquelle a été établie la procuration. Par ailleurs,

Je suis donc heureux que la commission ait enrichi le texte par un certain nombre de dispositions. À cet égard, je mettrai l'accent sur plusieurs mesures permettant de faciliter le recours au vote par procuration.

notamment lorsqu'ils présentent une vulnérabilité physique ou qu'ils ont été exposés au Covid-19. Un plus grand nombre de procurations doivent pouvoir être établies au domicile des électeurs et dans les hébergements collectifs, notamment au sein Je me réjouis également de l'adoption de deux dispositions visant à sécuriser les opérations de vote : la mise à disposition d'équipements de protection adaptés non seulement pour les électeurs qui n'en ont pas, mais également pour les personnes participant aux opérations électorales, et un meilleur encadrement de l'organisation du dépouillement. Chaque président de bureau de vote pourra en effet déterminer le nombre de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, en fonction des consignes sanitaires et de la superficie des locaux. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, 16,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 28 juin prochain, dans 4 857 communes, dont 1 442 communes de 1 000 habitants plus. Compte tenu de l'épidémie de Covid-19, ce scrutin implique de prendre un certain nombre de précautions. Cette proposition de loi permet, de manière très pragmatique, de renforcer la sécurité sanitaire dans tous les bureaux de vote. Les membres du groupe Les Indépendants partagent cet objectif et soutiennent sans réserve cette démarche.

et prolongeant le mandat des maires sortants. Si cette situation incongrue a été parfois compliquée dans certaines communes, elle a montré une fois de plus, et d'une manière très la solidité et le sens de la responsabilité des élus locaux. Les maires ont fait face avec détermination, courage et efficacité. Aujourd'hui encore,

La décision d'organiser le second tour des élections municipales le 28 juin prochain est sans doute pertinente, malgré des conditions de campagne difficiles, car la France doit revenir à la vie très rapidement. Pour cela, la gouvernance des collectivités doit être stabilisée, sécurisée, car d'autres coups de tonnerre nous attendent. En outre, les collectivités sont les acteurs indispensables de la relance économique.

s'impose naturellement. Nous adhérons donc totalement à la proposition de mise à disposition d'équipements de protection pour ces deux catégories de personnes, dans les 4 857 communes de France concernées par le second tour. Les collectivités ont dû et ont su pallier l'insuffisance des protections sanitaires, mais on ne peut aujourd'hui exiger d'elles qu'elles assument ce coût supplémentaire, qui relève de la vie démocratique. Il appartient donc à l'État de le financer. Le second défi, qui n'est pas le moindre, est démocratique. L'élection municipale est en général un scrutin au taux de participation significatif. de mars dernier, l'abstention a atteint plus de 52 % des inscrits, soit une hausse de près de 19 points par rapport à 2014. Nous devons aujourd'hui permettre au maximum des 16,5 millions d'électeurs appelés aux urnes le 28 juin d'exercer ce droit sacré qu'est le droit de vote. Les rassurer sur le risque sanitaire est indispensable, mais notre devoir est aussi de faciliter l'exercice de ce droit

saurait ! Quand des temps plus sereins seront revenus, il conviendra de réfléchir de manière plus large et plus approfondie à tous les dispositifs qui favorisent le vote et à leur sécurité. Si nous partageons la volonté d'encourager l'expression démocratique par le vote, il vous appartient d'être offensif quant à la mobilisation effective des autorités compétentes pour établir les procurations,

depuis le début de la crise, le Sénat n'a jamais failli à sa responsabilité, mes collègues l'ont rappelé : il a donné au Gouvernement des moyens exceptionnels, se délestant parfois même de certaines de ses prérogatives de législateur.

en permettant la prospérité rapide de cette proposition de loi en intelligence et en coopération avec le Sénat. La démocratie ne peut souffrir lenteur ou indifférence, en état d'urgence, car, après l'heure, ce n'est plus l'heure

Cette méthode, assez peu commune, répond à l'urgence de la tenue du prochain scrutin municipal prévu le 28 juin prochain, sous réserve d'un avis du conseil scientifique. Il s'agit donc de faire une bouture, en espérant que le greffon puisse prospérer dans le premier texte,

en étendant le recours aux procurations et en sécurisant l'organisation du scrutin pour les presque 17 millions d'électeurs des 4 857 communes concernées.

l'abstention aux élections municipales est un phénomène qui se développe dans le temps. L'élection locale n'échappe plus à la tendance globale à la désaffection à l'égard de la participation politique. Dans les années 1990, la participation aux municipales est passée sous la barre des 80 % ; dans les années 2000, elle s'est établie à moins de 70 %. Nous pensions avoir atteint un taux plancher en 2014, avec une participation de 63,5 %, et cela en dépit de l'attachement des Français à leur maire et à leur commune. La réponse abstentionniste est un mouvement de fond, symptôme d'un malaise de la représentation politique. Toutefois, l'effondrement de la participation du 15 mars dernier a une tout autre cause

le premier tour a eu lieu alors que l'on savait pertinemment que le second ne pourrait être organisé. Résultat, la participation s'est établie à moins de 45 %, chutant d'à peu près vingt points. Pour la première fois depuis le début de la V République, moins de la moitié des Français inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour une élection municipale. Dans un pays comme le nôtre, qui est viscéralement attaché au fait majoritaire, une participation en deçà des 50 % est très symbolique. Selon l'enquête Ipsos-Cevipof des 16 et 17 mars 2020, quelque 57 % des répondants qui n'ont pas participé au scrutin indiquaient ne pas l'avoir fait à cause du coronavirus. Cette abstention a été fortement différentielle. Toujours selon cette enquête, la proportion d'abstentionnistes a crû en fonction de l'âge : de 32 % parmi les 18-24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. 48 % des abstentionnistes des communes rurales ont invoqué le coronavirus, ce taux était de près de 70 % dans les communes urbaines. On peut donc en conclure que, d'une certaine façon, le scrutin du 15 mars dernier a été lui aussi infecté par le coronavirus.

auraient souhaité un report des élections. Par ailleurs, une autre enquête révèle que seul un tiers des électeurs concernés se disent prêts à se déplacer. L'organisation du scrutin ne fait donc pas consensus,

L'élection est coupée en deux, et il faut garantir le jeu démocratique lors d'un scrutin qui n'est vraiment pas comme les autres. Le conseil scientifique a invité à limiter les contacts pendant les campagnes et a énuméré des recommandations ; nous les partageons, elles sont reprises dans ce texte. Par ailleurs, des dispositions dérogatoires sont proposées s'agissant des opérations de vote. Elles peuvent se heurter aux standards électoraux qui qui font que la stabilité doit prévaloir. Je crois néanmoins que, dans la période que nous vivons, nous devons savoir faire preuve d'une certaine plasticité. Le texte de la commission propose d'étendre le recours aux procurations aux citoyens qui ne peuvent se rendre jusqu'à leur bureau de vote. L'élargissement du vivier des mandataires prévu par la loi Engagement et proximité est anticipé. Pourquoi pas ? C'est une bonne chose. Pourquoi s'arrêter là ? Nous défendrons des amendements visant à compléter cette mesure. Nous avons aussi conscience que ces dispositions nécessiteront une mobilisation des services de l'État comme des communes.

Là encore, ce n'est pas une solution parfaite, mais cela pourrait rassurer les électeurs. Si les estimations en matière de participation se vérifiaient, ce serait un problème non seulement pour le système politique, mais aussi pour les élus qui sont d'autant plus légitimes que la participation est forte.

nous pensons que la démocratie n'a pas de prix et nous devons la faire vivre, comme diraient certains, « quoi qu'il en coûte

Bien évidemment, ce texte est le produit d'un contexte très particulier, celui de la crise du Covid-19 et du report du second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines. Je rappelle que pas moins de 16,5 millions d'électeurs seront ainsi appelés aux urnes le 28 juin prochain dans quelque 4 857 communes, et ce dans un contexte sanitaire totalement inédit. Cela nécessite naturellement une organisation particulière du scrutin, qui implique de prendre un certain nombre de précautions sanitaires- c'est notamment ce qu'a préconisé le conseil scientifique dans son avis du 18 mai dernier. Il est donc particulièrement important de veiller à sa consolidation et à sa sécurité sanitaire dans tous les bureaux de vote. Dans cette perspective, je salue les travaux de la commission des lois, largement alimentés, il est vrai, par la proposition de loi déposée par nos collègues Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille, qui visait à mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales du mois de juin 2020. Ces travaux se sont concentrés sur deux axes prioritaires la sécurisation des conditions d'organisation du scrutin et la généralisation du recours aux procurations, en particulier pour les électeurs susceptibles de rencontrer des difficultés à se rendre dans les bureaux de vote. Ces deux points relèvent à la fois d'un enjeu de santé publique et d'un enjeu démocratique dont nous ne saurions nous affranchir, compte tenu de l'importance du vote. du vote. Je rappelle que le taux d'abstention a atteint plus de 55 % des inscrits lors du premier tour, soit une hausse de 18,8 points par rapport au scrutin de 2014. En ce qui concerne l'extension du recours aux procurations, le texte que nous examinons vise avant tout à garantir une meilleure information du mandataire d'une procuration, afin de s'assurer qu'il se rende au bureau de vote en lieu et place du mandant. En effet, la proposition de loi initiale vise à améliorer l'information du mandataire, en précisant qu'il est informé de la demande d'établissement de la procuration et des conditions d'organisation du vote. je rejoins l'initiative de Cédric Perrin de proposer un envoi électronique à l'adresse du mandataire, qui serait remplacé par courrier postal en l'absence d'accès à un moyen de communication dématérialisée.

lequel doit demeurer un geste démocratique essentiel et physique. Nous avons également proposé en commission qu'un même mandataire puisse recevoir deux procurations, afin de lui permettre de disposer d'une procuration supplémentaire établie sur le territoire national. Nous avons également assoupli la procédure afin de faciliter les procurations pour la famille proche, puisque, à titre dérogatoire un électeur pourra disposer d'une procuration dans une autre commune, mais uniquement pour voter au nom d'un ascendant, d'un descendant, de son frère ou de sa soeur. Enfin, je rejoins l'esprit de cette proposition de loi, qui est de protéger nos citoyens les plus fragiles en consacrant un droit pour certains électeurs d'établir leur procuration à domicile, notamment lorsque ces derniers risquent de développer une forme grave du Covid-19 ou qu'ils sont mis en quarantaine dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il me paraît cohérent d'étendre cette procédure au retrait des procurations. Dans cette perspective, si nous aidons une personne âgée à établir sa procuration, il faut également l'aider à la retirer si elle le souhaite. Par ailleurs, cette proposition de loi s'attache à sécuriser les opérations de vote. Il s'agit de préciser dans la loi que les équipements de protection tels que des masques devront être mis à la disposition des électeurs et de toutes les personnes qui participent aux opérations de vote- président de bureau, assesseurs, délégués du candidat, scrutateurs du dépouillement et agents communaux. Il semble plus que cohérent que cette dépense revienne à l'État, au même titre que les autres dépenses liées à l'organisation du scrutin. La stratégie sous-jacente de ce texte impliquera une grande mobilisation de la part du Gouvernement. Il incombera tout d'abord à ce dernier d'organiser un véritable service public des procurations. Il sera par ailleurs tenu de mobiliser les moyens nécessaires afin de permettre aux électeurs les plus fragiles d'exercer leur droit de vote. En effet, comment les collectivités pourraient-elles assumer, elles seules, la responsabilité de la sécurité sanitaire des opérations de vote ? En particulier, il ne saurait y avoir une sécurisation sanitaire des opérations de vote sans prendre en compte la question du dépouillement,

Finalement, elle ne faisait que rappeler la tradition républicaine de ne pas changer le droit électoral dans l'année précédant un scrutin, tradition consacrée dans la loi du 2 décembre 2019, sur l'initiative d'Alain Richard. Bien entendu, ce que la loi peut faire, elle peut aussi le défaire.

du droit électoral est une condition de la bonne information des électeurs et du bon fonctionnement de l'administration, ces deux éléments étant des préalables indispensables à la sincérité d'un scrutin. Aussi, faisons preuve de prudence, cette dernière étant d'autant plus nécessaire que la loi du 23 mars 2020, qui ne prévoit pas plus de trois mois entre les deux tours de scrutin de la même élection, pose des questions inédites en matière d'égalité et de sincérité du scrutin

entendu à mon compte les observations sur un second tour de scrutin où il sera possible de voter, mais pas vraiment de faire campagne, en tout cas de manière traditionnelle ; il n'est qu'à lire le rapport du conseil scientifique ou qu'à entendre les craintes de nombre de nos compatriotes sur les risques sanitaires pris par les électeurs, mais aussi, et peut-être surtout, par tous ceux qui tiendront les bureaux de vote. L'abstention que cela pourrait provoquer est problématique. Je comprends donc la démarche de plusieurs de nos collègues. Mais compte tenu des principes affirmés précédemment, modifier des règles en cours de route ne serait probablement pas convenable, surtout s'il s'agissait de mettre en oeuvre un dispositif de vote par correspondance qui n'est plus utilisé depuis longtemps, qui ne participe plus de notre tradition républicaine et qui, lorsque lorsque nous l'utilisions, fut vecteur de nombreuses contestations, qui ont conduit à l'abandonner. Enfin, alors qu'il est probable que cette proposition de loi ne puisse être adoptée avant le scrutin du 28 juin je crains qu'elle ne participe à brouiller la compréhension de ce scrutin et de ses règles par nos concitoyens, au lieu d'apporter une réponse réelle à l'enjeu majeur et essentiel de la participation. La parole

célébrant le rituel républicain du vote, Victor Hugo écrivait en 1850 : « Il y a dans l'année un jour où le plus imperceptible citoyen participe à la vie immense du pays tout entier, où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui l'âme de la patrie ! » Les jours d'élection demeurent le moment le plus emblématique de l'exercice de la citoyenneté. Ils s'accompagnent, au sein des bureaux de vote, d'un rituel formalisé, associé au matériel, familier à l'électeur : les bulletins, l'isoloir et l'urne transparente. Plusieurs dispositions de la partie législative du code électoral ont constitué lors de leur adoption de véritables innovations. Elles tendaient à garantir la confiance que les citoyens placent dans les opérations électorales, condition de la légitimité des résultats du scrutin. La Constitution elle-même veille sur ce pacte républicain. Le juge de l'élection s'assure de l'égalité des citoyens, du secret du vote et de la sincérité du scrutin. Lorsque la législation électorale est modifiée, le juge constitutionnel contrôle sa conformité à ces mêmes principes. Le principe de secret du vote exige que l'électeur émette son suffrage hors de tout regard extérieur, condition de sa liberté. La suppression du vote par correspondance en 1975 et l'installation de machines à voter, d'abord mécaniques, puis électroniques, ou encore les essais de vote par internet ont élargi les possibilités, mais avec beaucoup de réserves.

par internet me paraît une absurdité. » Devant une telle insistance, ce texte me donne l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Si les présentes élections revêtent une particularité sanitaire qui ne doit cependant pas empêcher la volonté et la possibilité de chacun de voter, il n'est pas possible de s'avancer sur le vote électronique sans en connaître les dangers.

Ce document en exposait les mérites et les risques. Nous nous étions alors prononcés pour le maintien de la situation actuelle : poursuite du vote par internet seulement pour les Français établis à l'étranger, à l'occasion des élections en matière de vote à distance, la sécurité est d'autant plus délicate à garantir que la puissance publique n'a aucune prise ou aucun moyen de contrôle sur le terminal qui sert à l'électeur pour voter. Celui-ci choisit librement le terminal de vote, le plus souvent un ordinateur personnel. d'information (Anssi), les moyens pour parer à tous les risques informatiques sont hors de prix pour un simple particulier. Ce risque est d'autant plus fort que, selon les électeurs, les terminaux varient, de même que les logiciels et les navigateurs. En matière de secret, l'absence d'un cadre formel comme le passage dans l'isoloir n'assure pas les conditions garantissant le caractère non public du vote. L'électeur peut voter devant son ordinateur sous le regard, donc sous la pression plus ou moins forte d'un tiers. Tel le cas des personnes frappées d'illectronisme, soit par l'âge, soit par manque de formation.

ne se sont pas développées. Il n'est qu'à voir les élections américaines de la fin de l'année 2016 et la suspicion à l'égard de la Russie, accusée d'avoir mené des attaques et des interférences au cours de la campagne qui a précédé ce résultat. Cette situation a amené le ministère de l'intérieur à exclure, au mois de mars 2017, le recours au vote électronique pour les citoyens français de l'étranger

Enfin, selon le spécialiste du droit électoral Romain Rambaud, « on ne peut mettre en place » le vote électronique « un mois seulement avant le scrutin, en raison du principe de stabilité du droit électoral ». Pour ce scrutin municipal de second tour, il n'est évidemment pas possible, comme certains l'ont réclamé haut et fort, de déployer un système sécurisé, facile d'utilisation et résilient, déjà perfectible pour un scrutin national. C'est inenvisageable pour près de 5 000 communes et 16,5 millions d'électeurs. Malgré le temps réduit qui restera au Gouvernement pour organiser ce que le président de la commission a justement nommé le « service public des procurations »,

que ce second tour des élections municipales, le 28 juin prochain, puisse avoir lieu dans des conditions permettant de faciliter la participation au vote de nos concitoyens. Monsieur le secrétaire d'État, si vous avez

fut encore le cas récemment sur la durée des campagnes électorales ou sur les caractéristiques des bulletins de vote, pour interdire par exemple des photographies sur les bulletins de vote ou la représentation d'un animal. des dispositions d'ordre réglementaire, mais le Parlement se reconnaît une petite liberté dans l'appréciation de ce qui est réglementaire ou de ce qui ne l'est pas, étant entendu que les termes de l'article 34 de la Constitution sont assez

également de la loi. Il nous semble que, pour l'essentiel, les dispositions que nous vous proposons peuvent figurer, sans préjudice pour l'étendue du pouvoir réglementaire, dans un texte législatif. Par ailleurs, si je comprends bien, le problème, c'est le choix du texte législatif.

pas rappelé -d'annuler le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, etc., et d'organiser un nouveau scrutin, qui pourrait se dérouler jusqu'au 31 janvier 2021 pour pourvoir les sièges de conseillers municipaux qui n'ont pas été définitivement attribués le 15 mars dernier. Dois-je comprendre

Qui plus est, je ne suis pas du tout certain que ce texte pourra aboutir plus rapidement que celui que nous vous avons présenté, quand bien même vous auriez décidé d'engager la procédure accélérée. Vous le savez, il est bien rare

créant l'état d'urgence sanitaire et en cinq jours la loi le prorogeant. À partir du moment où cette coopération entre le Gouvernement et le Parlement, notamment le Sénat de la République, s'était enclenchée, nous avons eu l'illusion- oserais-je dire la naïveté ? -de penser que, pour des raisons d'intérêt supérieur, le Gouvernement utiliserait non pas un vecteur inapproprié et qui n'aboutira pas à temps, mais un vecteur qui a toutes les chances

Herzog. Cet amendement a pour objet d'interdire l'utilisation des listes d'émargement du premier tour pour démarcher les électeurs. Cette mesure est d'autant plus importante que les maires sortants ont accès aux listes d'émargement et sont les seuls à pouvoir utiliser ces documents pour solliciter des procurations.

Quel est l'avis de la commission ? le texte de la commission constitue déjà une avancée non négligeable pour les électeurs. En outre, la plupart des Français établis hors de France sont aujourd'hui inscrits sur la liste électorale consulaire et, depuis 2016, ils ne peuvent plus être inscrits de manière

aux membres de la famille proche le vivier des personnes non électrices de la commune susceptibles de recevoir procuration.

C'est la raison pour laquelle nous avons voulu limiter à une dérogation pour les membres de la famille proche la possibilité de détenir une procuration pour une personne non électrice

en raison de cette difficulté pratique que nous n'avons pas donné un avis favorable à votre premier amendement. En revanche, la commission, après en avoir longuement délibéré ce matin, a accepté de modifier le périmètre de la famille proche. Il arrive en effet que des conjoints,

qu'une personne âgée vivant en maison de retraite médicalisée appelle la gendarmerie pour donner une procuration sans raison

opérationnalité le droit de la personne à donner procuration. C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'État, nous tenons à donner une portée législative

le fait que les procurations restent valables peut poser de nouvelles difficultés. Certains mandants qui souhaitent aller voter devront se déplacer pour faire savoir qu'ils renoncent à leur procuration. De plus, les services compétents peuvent être amenés à

il faut proposer le maximum de dispositifs pour permettre à nos concitoyens de toutes conditions et de tous âges, pour autant qu'ils soient en âge de voter, d'exercer leur droit de vote.

Si nous le mettons en oeuvre pour les élections du 28 juin, nous aurons une petite chance de réacclimater une procédure qui présente pour l'électeur un double avantage : il n'a à confier son choix à personne et il dispose d'un équivalent de l'isoloir pour exprimer secrètement son choix.

La première porte sur le matériel de vote par correspondance : celui-ci est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième mercredi qui précède le scrutin-il va donc falloir aller vite. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification et une enveloppe électorale. Pour permettre le contrôle de son identité- c'est la deuxième garantie -, l'électeur signe l'enveloppe d'identification et y insère une copie d'une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile. Son pli est transmis, non pas à la mairie, mais au tribunal judiciaire, soit par voie postale, soit par le gendarme ou le policier assermenté. Troisième garantie : dans l'attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d'instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d'ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre.

sont compétents pour établir les procurations. Quatrième garantie : à la clôture du bureau de vote, le président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d'émargement et introduisent l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'urne, après s'être assurés que l'électeur concerné n'a pas déjà voté.

au temps de mise en place de la logistique qu'impose le vote par correspondance, notamment l'acheminement des enveloppes, qui,

Deuxièmement, ce vote est neutre du point de vue politique. Il a été prouvé qu'il ne bénéficie pas plus à une formation qu'à une autre.

après le vote des ides de mars, vous nous proposez le vote par correspondance aux calendes grecques, ces calendes qui n'existent pas

que la distribution de masques, que le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à prendre à sa charge, a un impact sur le vote, puisqu'elle permet de rassurer un certain nombre de personnes qui n'en auraient pas chez

pour permettre l'expression du suffrage universel avec un minimum d'abstention le 28 juin prochain. M. Perrin est l'auteur de la proposition de loi sans laquelle nous ne serions pas réunis ici. J'ai donc beaucoup de scrupules à lui demander de retirer son amendement. Je le fais néanmoins, sans excès de conviction. Je le laisse juge de ce qu'il convient de faire dans l'intérêt

L'accès à l'isoloir et la normalisation des outils du vote ont eu un rôle essentiel dans notre démocratie électorale. Pour autant,